de l'ordonnance du 29 janvier 2016, relatifs aux conditions de modification d'un contrat en cours et aux conditions d'indemnisation d'un concessionnaire. La modification proposée consiste à créer un parallélisme avec la disposition prévue par l'article 21 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

du Gouvernement ? L'amendement tend à appliquer les règles des concessions en ce qui concerne la modification des contrats en cours et l'indemnisation des cocontractants pour les contrats de service public qu'Île-de-France Mobilités va mettre en concurrence en vue de l'exploitation des lignes

B à court terme. Nous pensons, pour notre part, que l'amélioration de la desserte de l'aéroport doit s'effectuer dans le cadre du service public et profiter ainsi aux Franciliens des villes populaires, comme La Courneuve, Aubervilliers, Le Blanc-Mesnil, Drancy, Aulnay-sous-Bois, etc.

et nous le répétons : faire le choix du Charles-de-Gaulle Express, c'est renoncer à améliorer les conditions de transport des usagers du quotidien. En ce sens, ce projet est symbolique d'une conception des transports publics aux antipodes de la nôtre, à savoir répondre aux besoins du plus grand nombre en desservant au plus près les territoires. Au travers de cet amendement, nous souhaitons donner la priorité aux transports des Franciliens. semble impératif, dans cet esprit, de mettre un terme à un projet dispendieux et inégalitaire, sans justification économique, environnementale ou sociale, un projet qui suscite une véritable opposition des usagers et des élus

un seul exemple : les bagages abandonnés par les usagers de Roissy causent de nombreux arrêts et retards sur la ligne. Sur le principe, l'idée de créer une liaison dédiée entre la capitale et l'aéroport était donc excellente, des transports du quotidien que du rayonnement et de l'attractivité de la métropole parisienne. Malheureusement, le projet actuel ne prévoit plus de liaison dédiée : les questions de calendrier liées à l'accueil des jeux Olympiques ont eu raison de la bonne idée initiale Charles-de-Gaulle Express, avec son tracé actuel, empiètera, en phase de travaux comme en phase d'exploitation, sur les tronçons déjà saturés et dysfonctionnels du faisceau nord francilien. Jusqu'à présent, la forte mobilisation des usagers et des associations n'a pas permis d'obtenir de modification du projet, mais chacun sent bien que cette situation n'est pas tenable. Nombreux sont les acteurs qui disent tout bas ce que personne ne veut assumer tout haut : le projet actuel et son calendrier sont déraisonnables. Cela rappelle d'ailleurs ce que l'on entend dire du projet Grand Paris Express en général ... Il y a deux jours, le 26 mars, le journal révélait même que SNCF Réseau pousse au report d'au moins dix-huit mois du projet, pour éviter un impact trop fort sur les trains du quotidien pendant les travaux. Madame la ministre, vous êtes très engagée pour les transports du quotidien, or tout porte à croire que le projet du Charles-de-Gaulle Express va les pénaliser très lourdement. Il est nécessaire de le revoir.

en Île-de-France, avec un contrat de plan de 7,6 milliards d'euros et le projet du Grand Paris Express, qui représente un investissement de 35 milliards d'euros. Les transports du quotidien sont donc bien la priorité du Gouvernement, et ils le resteront ! Dans ce contexte, je voudrais rappeler que le projet du CDG Express ne suppose aucune subvention publique : il sera financé en totalité par les passagers du transport aérien et les clients du CDG Express. Au sein de

Cette façon de légiférer ne respecte pas les droits des parlementaires que nous sommes. Nous voulons pouvoir disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à la réflexion. Nous voulons également obtenir de votre part l'assurance que ces dispositions sont le fruit d'un véritable dialogue social avec les organisations syndicales. Pour en finir avec la forme, nous regrettons que plusieurs de nos amendements à cet article

Ils expriment notre volonté de sécuriser les parcours des agents du service public, qui ont, lors de leur embauche, bénéficié d'un certain nombre d'avantages, notamment la garantie de l'emploi. Nous espérons que nos échanges permettront de réelles avancées pour eux et pour tous les agents des transports publics, grâce à une réelle harmonisation

territorialisé nous paraît opportune, car cela permet de prendre en compte les spécificités de certaines zones géographiques. Nous soulignons l'esprit de

nos collègues du groupe CRCE. Il est évident que le volet social de cette ouverture à la concurrence est un sujet extrêmement sensible. Ces transferts pourront constituer un véritable bouleversement pour les salariés qui perdront le bénéfice du statut RATP et verront leurs conditions de travail modifiées. Nous serons

Dix ans après, il était plus que temps de définir le cadre social applicable à cette ouverture à la concurrence ; c'est ce que nous faisons. Je considère qu'il est de notre responsabilité d'agir pour que ce processus se déroule dans de bonnes conditions, permettant de concilier la continuité du service et le libre choix de l'opérateur par l'autorité organisatrice, mais surtout d'assurer la mise en place de garanties sociales de haut niveau pour les salariés. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, les agents de la RATP affectés au transport par bus sont en effet susceptibles de changer d'employeur. Le changement d'employeur n'est jamais neutre, pour les agents issus de la RATP,

les conditions de circulation et d'exploitation des réseaux de bus dans la zone dense urbaine francilienne sont soumises à des contraintes qui ne se retrouvent dans aucun autre réseau. Là encore, cela n'aurait pas de sens de faire table rase du passé et de prétendre appliquer à Paris et au coeur de l'Île-de-France ce qui se fait ailleurs. Les conséquences en seraient désastreuses, notamment pour la continuité de service.

la cinquantaine de réunions de concertation qui se sont tenues avec les partenaires sociaux de la RATP et de la branche du transport public, en y associant l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilités. Je voudrais saluer l'esprit de responsabilité

qui repose, d'une part, pour les conducteurs de bus, sur la mise en place d'un cadre social adapté à un territoire spécifique, avec des règles spécifiques en matière de temps de travail et de repos, et, d'autre part, pour l'ensemble des salariés affectés à ces activités de transport par bus, sur un dispositif définissant les modalités de transfert des salariés et les garanties apportées à ceux-ci. Par ailleurs, les concertations se poursuivent pour finaliser le cadre social. D'autres amendements devront donc sans doute être introduits à l'Assemblée nationale. nationale. Il s'agira notamment de préciser les conséquences du refus de transfert pour les salariés. C'est ce point particulier qui reste à définir s'agissant des salariés de la RATP. Je voudrais aussi souligner, en réponse

la commission et son rapporteur ont été en lien régulier avec le Gouvernement sur ces dispositions qui revêtent un caractère sensible. Je salue cette méthode de travail, et je remercie Mme la ministre de m'avoir associé régulièrement à ses réflexions.

Notre rôle est de sécuriser les droits des salariés et de créer les conditions requises pour garantir la continuité et la qualité du service, dans l'intérêt de tous les acteurs et des usagers. Je donnerai en conséquence,

objet de garantir que ce transfert se fera sur la base du volontariat. Il nous paraît en effet essentiel de laisser aux salariés la possibilité de s'exprimer sur le sort de leur contrat de travail, dans la mesure où l'on peut craindre que l'ouverture à la concurrence

Les salariés ne sont pas de simples outils de production transférables à volonté à l'entreprise qui remporte le marché public. Les changements successifs d'employeur, combinés à la mise en concurrence, pouvant entraîner une dégradation des conditions de travail, ils doivent avoir leur mot à dire, particulier lorsque leur contrat de travail fait l'objet d'une modification aussi importante qu'un changement d'employeur, lequel emporte nécessairement des conséquences sur les modalités d'exécution du contrat comme sur la qualité des conditions de travail.

Il pose le principe d'une information claire et précise des salariés tout au long du processus d'ouverture à la concurrence et vise à déterminer le nombre de salariés à transférer pour faire fonctionner le service, ainsi que les critères de désignation des salariés dont le contrat de travail sera effectivement transféré.

faire toute leur carrière à la RATP. Dans un contexte d'ouverture à la concurrence, il n'est pas envisageable de ne pas leur garantir certains droits spécifiques. À ce titre, tous les salariés bénéficieront, notamment au moment du transfert, d'une garantie de rémunération et du maintien de leurs accords collectifs pendant une durée de quinze mois maximum, ainsi que de l'accès au centre de soins de la RATP et, pendant douze mois, à ses activités sociales et culturelles. Quant aux salariés sous statut, ils bénéficieront de la portabilité, de la garantie de l'emploi et du régime spécial de retraite, qui sont des éléments structurants de leur statut.

est à Mme la ministre. Au travers de cet amendement, il s'agit de garantir la continuité du service et la sécurité des circulations au sein d'un périmètre géographique parisien et francilien caractérisé, comme nous le savons tous, par des conditions d'exploitation des bus que l'on ne rencontre pas ailleurs. Cet amendement tend à compléter la liste des dérogations possibles à certaines dispositions législatives du code du travail en matière de durée du travail, de congés et de repos des conducteurs opérant à l'intérieur de ce périmètre. L'amendement vise non pas à fixer le contenu des règles applicables, mais à autoriser le pouvoir réglementaire à le faire en vue de définir un cadre social territorialisé, qui s'appuiera sur le décret du 14 février 2000 sur la durée de travail dans les entreprises de transport public urbain et, si les partenaires sociaux de la branche en décident ainsi, sur un avenant territorial à la convention collective du transport public urbain. Continuant de s'appliquer en l'état aux salariés de la branche du transport public urbain, le décret de 2000 sera complété par une annexe définissant les règles spécifiques applicables en matière de durée du travail et de repos aux conducteurs de bus opérant sur des lignes dont le parcours est majoritairement effectué dans la zone urbaine dense francilienne. Ces règles spécifiques tiendront compte des conditions particulières d'exploitation dans cette zone et pourront notamment porter sur le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, la réduction du repos quotidien, l'adaptation du délai de prévenance en cas de changement d'horaire par l'employeur, ainsi que sur les contreparties associées en matière de repos, de jours de congé et de modalités de fixation des jours fériés chômés qui sont nécessaires pour garantir la sécurité des circulations. L'amendement n° 205, présenté par Mme Assassi,

pour l'offre de transport public, car il amène ces agents à développer un sens aigu du service public et de l'intérêt général, indispensable notamment en temps de crise ou lors d'événements majeurs. Nous demandons donc la suppression de ces dispositions, dont l'application généralisée la fin du statut spécifique de la RATP et son remplacement par une convention collective valable pour l'ensemble des agents du réseau de bus.

vise à préciser que la convention collective du transport public urbain, qui n'a pas été négociée en vue de s'appliquer aux conducteurs de bus intervenant dans la zone RATP, ne s'applique pas aux agents de la RATP, en cohérence avec le cadre spécifique qu'il est proposé de créer. Cet amendement vise à garantir l'application du cadre social territorialisé à tous les conducteurs de bus qui interviennent dans le périmètre de la zone dense urbaine, quelle que soit la convention collective applicable à leur employeur.

vous souhaitez introduire la notion de volontariat, sans doute par analogie avec ce qui avait été prévu pour les salariés de la SNCF. En réalité, les deux situations sont très différentes : à la SNCF, l'organisation du travail fait que certains

vous souhaitez préciser que le transfert se fera dans le respect des métiers et de l'organisation collective de travail. S'agissant des métiers, cet amendement est satisfait, puisqu'il est précisé dans le texte que les salariés transférés seront désignés par catégories d'emploi, et donc dans le respect des spécificités de leur métier. En revanche, si vous souhaitez

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement n° 600 rectifié, consistant à privilégier la négociation collective plutôt que la voie réglementaire pour fixer les règles relatives à la durée du travail et au repos applicables aux salariés de la RATP.

Quel est l'avis du Gouvernement ? De manière générale, je privilégie la négociation collective, mais, en l'occurrence, compte tenu de la nécessité de fixer rapidement le cadre applicable à l'ensemble des acteurs concernés par l'ouverture à la concurrence et, par ailleurs, de définir un socle minimum de garanties pour les salariés qui s'imposeront à tous, il est nécessaire de passer par un décret. Cela ne prive pas les partenaires sociaux de leurs prérogatives, puisqu'il leur sera ensuite possible de négocier au niveau de la branche du transport public urbain, de même que dans les entreprises, des dispositions venant compléter ou préciser le décret.

Monsieur le rapporteur, je compte beaucoup sur vous pour cet amendement, qui vise à permettre à Île-de-France Mobilités d'émettre un avis consultatif avant la fixation par l'État du cadre réglementaire délimitant le périmètre géographique des communes présentant des contraintes spécifiques d'exploitation. Il semble en effet souhaitable que les collectivités territoriales et l'autorité organisatrice soient consultées avant la définition de ce périmètre.

fragiliserait le CST, qui permet d'imposer des contraintes particulières aux salariés, au bénéfice de la collectivité. Je souhaite le retrait de cet n° 974 rectifié ne me semble pas nécessaire : la durée légale du travail visée à l'article L. 3121-27 du code du travail ne constitue pas une obligation de travailler 35 heures, mais définit le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

de tenir compte des contraintes d'exploitation propres à certaines communes. Par ailleurs, l'article 39 a bien pour objet de placer les salariés concourant à l'exploitation des bus dans le cadre du régime du code du travail. Je considère donc que cet amendement est

De nombreux services sont concernés dans un délai court, avec une seule autorité organisatrice chargée de conduire le processus. En conséquence, la loi doit permettre de prendre en compte les éventuels délais de procédure qui aboutiraient à différer, de manière limitée, le changement effectif d'attributaire du contrat.

pour les conducteurs éludant de manière habituelle le paiement du péage. Les trois

relatives au délit d'habitude avec celle de l'article L. 121-2 du code de la route, qui fixe les principes de la responsabilité pénale en cas d'infraction à la réglementation sur l'acquittement des péages.

L'esprit général du texte est toutefois préservé : il y a toujours une incitation à éteindre rapidement la procédure par la minoration de l'indemnité forfaitaire, et l'échelle des sanctions est durcie, avec la création d'une amende de 7 500 euros, la peine de prison ayant été

la mesure proposée s'appliquerait à toutes les amendes forfaitaires majorées, ce qui nous paraît excessif. Cela enlèverait toute marge de manoeuvre au comptable public, alors que le dispositif actuel constitue une incitation pour les conducteurs non vertueux.

vise à revenir sur des dispositions adoptées en commission. Si nos collègues estiment que l'opposition obligatoire au transfert du certificat d'immatriculation pour les seules infractions liées au passage en flux libre est nécessaire pour accompagner indirectement la lutte contre la fraude, j'émettrai un avis

je souhaiterais qu'on en reste là. Madame la ministre- je le dis sans faire allusion à des dispositions dont nous avons débattu hier -, il faut que nous soyons pragmatiques. L'introduction du péage à flux libre est une bonne chose,

évaluent la perte potentielle liée à la mise en place du flux libre à environ 5 % du montant total des recettes actuelles. [ ...] Elles estiment ainsi que le déploiement de ce système pourrait représenter un manque à gagner de l'ordre de 500 millions d'euros par an à l'échelle nationale sur les 10 milliards de revenus des péages autoroutiers.

L'autoritarisme est contre-productif : les punitions trop sévères, infondées surtout, sont génératrices de phénomènes de fond extrêmement graves, notamment le non-consentement aux redevances et aux taxes.

car le dispositif de péage en permet avant tout la facturation, et non la perception du péage. Pour la seconde partie, dans la mesure où l'usager ne respecte pas le délai de post-paiement, il sera formellement considéré comme ayant R. 421-9 du code de la route, et une contravention sera dressée. Il ne paraît pas possible de superposer cette procédure à la transaction du concessionnaire. Je demande donc le retrait des amendements ; à défaut,

Malgré le constat largement partagé de l'erreur que fut leur privatisation, la majorité du Sénat a voté l'amendement de suppression

Comme si la puissance publique ne pouvait faire le choix de défendre ses intérêts stratégiques ... Bref, un consensus s'est dégagé pour attendre la fin des concessions ; peut-être, à ce moment-là, pourrons-nous examiner la possibilité d'une reprise.

nous pouvons partager votre préoccupation quant aux modalités de contractualisation. Toutefois, interdire globalement le recours à la concession n'est pas souhaitable : c'est un mode de réalisation de travaux d'exploitation qui permet à la personne publique de ne pas supporter des risques économiques et financiers, tout en s'appuyant sur l'expérience d'entreprises solidement établies. Avec une bonne négociation, la concession peut être un choix rationnel et adapté à tout type de projets. L'avis est donc défavorable.

titre personnel. Pour autant, il ne faut pas condamner les montages concessifs, qui ont permis de développer un réseau de près de 10 000 kilomètres, très utile y compris en termes d'aménagement et de développement de notre territoire. Ces procédures

En France, la question de la concurrence sur le marché aval des travaux s'est posée, en raison de l'appartenance de certaines sociétés d'autoroutes à des groupes de travaux publics. Le Parlement a donc souhaité encadrer spécifiquement ces marchés, mais le texte de loi n'a pas limité le domaine d'application de cet encadrement. Conformément à la directive, le périmètre d'application de l'encadrement des marchés devrait spécifiquement être adapté à l'enjeu particulier l'ayant motivé. Les autres contrats passés par les sociétés d'autoroutes ne présentant aucune particularité par rapport à ceux passés par d'autres délégataires, la situation actuelle est constitutive d'une rupture d'égalité devant la loi. Dans le cas concret des sociétés d'autoroutes, lors de l'analyse de leurs achats et des secteurs où interviennent les entreprises qui leur sont liées, le constat, évident, est que le seul type d'achats qui puisse éventuellement poser problème est celui des travaux commandés à des entreprises liées. D'une part, les sociétés d'autoroutes ne sont pas des acheteurs importants de fournitures et services, certainement pas au point de peser sur les marchés sur lesquels elles achètent des fournitures et services. Les entreprises qui leur sont liées ne sont d'ailleurs pas présentes sur ces marchés et n'y disposent à coup sûr pas d'une position importante. Il convient donc d'exclure de tout encadrement spécifique les achats de fournitures et services des sociétés d'autoroutes. Quel est l'avis de la commission

n'a pas encore eu le temps de publier le rapport quinquennal sur l'économie générale des concessions qu'elle doit remettre en application de l'article L. 122-9 du code de la voirie routière. Cette loi de 2015 conduit à renforcer la régulation du marché de l'autoroute concédée

doivent rester contrôlés par l'Arafer ; je pense, par exemple, aux marchés de maîtrise d'oeuvre. Je comprends bien votre souci de simplification,

proposez. Le code de la voirie routière prévoit d'ores et déjà des modulations horaires et environnementales, les modulations environnementales étant obligatoires pour les poids lourds. S'agissant des voies réservées pour le covoiturage ou les transports en commun, elles sont étudiées et contractualisées au cas par cas. Cette démarche n'est pas

n° 316 rectifié est retiré. Madame la ministre, mes chers collègues, je suis heureux de saluer la présence dans nos tribunes des auditrices et des auditeurs de la quatrième promotion de l'Institut du Sénat. l'initiative de notre ancien collègue Jean-Léonce Dupont, le bureau du Sénat avait décidé, en 2015, de mettre en oeuvre ce programme de formation, en vue de mieux faire connaître les modalités de fonctionnement et les enjeux de notre démocratie parlementaire à des personnalités d'horizons géographiques et professionnels très divers. auditeurs de cette quatrième promotion, qui sont issus des quatre coins de notre pays, représentent en effet toutes les sphères d'activité professionnelle : publique, économique, sociale, associative, syndicale ou encore universitaire. de leurs travaux, qui ont commencé il y a deux semaines et s'achèveront à la fin du mois de juin, ils rencontreront plusieurs de nos collègues sénateurs et des fonctionnaires du Sénat. En votre nom à tous, je leur souhaite une excellente session au Sénat, et je suis certain que, à l'issue de ces trois mois, ils pourront être les témoins privilégiés de la place essentielle de notre institution au sein de la V République et de la qualité du travail parlementaire.

l'automobiliste est la mauvaise variable d'ajustement. Un kilomètre d'autoroute gratuite constitue une charge de fonctionnement pour le ministère des finances. J'ai le cas en Lorraine : un kilomètre

et demi des concessions concernées. Mais aujourd'hui, le financement de tels adossements ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs des péages, ce que je conteste. je propose de réintroduire la possibilité de financer certains projets par un allongement raisonnable de la durée de la concession. Permettez-moi, madame la ministre, de prendre l'exemple, dans mon département de l'Hérault, du projet de liaison entre l'A 750 et

Aucune autre solution ne peut être sérieusement envisagée pour financer en totalité ce chaînon manquant entre l'A 750 et l'A 709 dans la métropole de Montpellier, sauf à créer une autoroute à péage,

Il serait tout à fait souhaitable qu'il y ait davantage de transparence. À cet égard, je me réjouis que le Conseil d'État ait enfin condamné l'État et les sociétés d'autoroutes à porter à la connaissance du public le contenu des contrats qui ont été signés en 2015. J'indique que, en tant que président de commission, j'avais écrit au Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, au ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, et à la ministre de l'écologie de l'époque, Mme

toujours plus gros et aux compétences de plus en plus larges. Elles ne sont pas étrangères à la lassitude et au désarroi des maires et de l'ensemble des élus municipaux. Pour les communautés urbaines et les métropoles, le transfert obligatoire de la compétence pour toutes les voiries s'est souvent opéré au prix d'un grand nombre de difficultés.

le rappelle, ce sont les communes qui, les attributions de compensation, financent ces travaux. En outre, il n'y a aucune recherche de concours financiers pour augmenter les recettes, aucune garantie que les travaux correspondent parfaitement aux attentes du maire et des usagers,

je propose d'établir une hiérarchisation des voiries, en distinguant les voiries d'intérêt communautaire, relevant de l'EPCI, et les voiries d'intérêt communal, relevant de la commune.

ce qui implique que les communautés urbaines et les métropoles exercent des compétences d'ultraproximité, dont l'entretien quotidien de la voirie, alors que ces EPCI devraient se concentrer sur la stratégie territoriale et les grands plans d'aménagement. Cela conduit ces EPCI à se détourner de leurs missions véritables et engendre un sentiment de dépossession des maires à l'égard de leurs administrés. En conséquence, cet amendement vise à restreindre la compétence de la communauté urbaine et de la métropole à la voirie principale déterminée d'intérêt communautaire ou métropolitain par l'organe délibérant. L'avis est favorable. Quel est

et le ministère des transports ont souhaité sécuriser le régime social et fiscal du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, spécifique à cette branche. Cet amendement permet de répondre à une attente forte de la profession.

transports routiers. D'après les informations qui ont été portées à notre connaissance, cette demande vient du fait qu'il existe parfois des divergences d'appréciation entre certaines Urssaf et les entreprises de transport sur les modalités de remboursement de ces frais.

du 20 février dernier, prolonge l'habilitation du Gouvernement à déterminer par voie d'ordonnance les conditions de négociation collective au sein de la branche ferroviaire, afin notamment de tirer les conséquences de l'éventuelle absence de conclusions de la convention collective de branche au 31 décembre 2019. En cohérence avec la position que nous avons défendue lors de l'examen du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire et notre refus de la fin du statut des cheminots au 1janvier 2020, nous ne souhaitons pas que soit prolongée l'habilitation à légiférer par ordonnance dans un domaine,

aux ordonnances en matière sociale. Il s'agit en effet, sous couvert de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l'absence de conclusion d'accords collectifs dans un délai déterminé, de créer les conditions juridiques permettant d'imposer aux salariés une nouvelle convention collective ou, pour le moins, d'en brandir la menace. La rédaction de cet article, qui permet au Gouvernement de tirer les conséquences de l'absence d'accords, est beaucoup trop vague à nos yeux et mériterait d'être précisée. Étant extrêmement attachés à la défense des droits des cheminots, qui sont le coeur du service public ferroviaire, nous ne souhaitons pas qu'une simple ordonnance puisse porter atteinte à des droits collectifs acquis. Nous appelons encore une fois le Gouvernement à revenir sur l'extinction du statut des cheminots. Quel commission ? Le prolongement de l'habilitation à légiférer par ordonnance pour sécuriser les négociations de la branche du transport ferroviaire, disposition que nous avions initialement adoptée dans la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, mais qui a expiré,

Mme la ministre.

de loi. Notre amendement vise à sécuriser la continuité des droits des salariés transférés à un nouvel attributaire d'un contrat de service public en cas de sous-traitance mise en place pour la réalisation de l'activité transférée et de transfert ultérieur des contrats de travail vers ce ou ces sous-traitants, que ceux-ci soient des entreprises filiales ou des entreprises tierces. Il s'agit d'assurer l'application pleine et entière des garanties données par la loi aux salariés

les réticences, voire les blocages, lors des transferts d'activités et des contrats de travail nécessaires à leur réalisation. C'est une condition directe de la continuité du service public lors des changements d'attributaire. Il s'agit en quelque sorte d'un amendement

la commission ? Il me semble que cet amendement est satisfait, car la loi pour un nouveau pacte ferroviaire dispose que les salariés transférés à une nouvelle entreprise bénéficient de certains droits garantis, y compris quand leur contrat de travail est ultérieurement transféré à une autre entité. Sous réserve des précisions que pourra nous apporter la ministre sur ce point, la commission émet un avis défavorable madame la ministre, mais sous réserve que le salarié reste couvert par les stipulations de la convention collective de la branche ferroviaire. Le cas de figure visé ici est, par exemple, celui de salariés chargés de la maintenance du matériel ferroviaire qui pourraient être

priorité à la mobilité volontaire des salariés dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, notamment négociation collective expressément prévue par la loi permettra de fixer les conditions dans lesquelles ce dispositif, prévu par le code du travail pour favoriser et faciliter des parcours professionnels interentreprises, pourra s'appliquer dans le cadre d'un changement d'attributaire d'un contrat de service public. Une telle disposition

le dispositif de transfert des salariés, sachant que le délai de six mois laissé à la négociation collective n'a pas permis de traiter le sujet. L'attractivité du volontariat s'en trouvera renforcée. La réussite du volontariat dans le cadre des changements d'attributaire est un facteur facilitant l'engagement des salariés dans ces évolutions et, par là même, le moyen d'éviter des blocages. C'est une condition directe de la continuité du service public lors des changements d'attributaire. Quel est l'avis de la commission

Mme la ministre.

paraît superflue, étant donné que, chaque année, la SNCF publie dans son rapport financier les éléments relatifs à la gestion du groupe et à sa situation financière, ce qui permet de mesurer d'éventuels écarts par rapport aux objectifs fixés par le contrat-cadre conclu avec l'État.

Ceux-ci, lorsqu'ils se mettent en grève, défendent leur outil de travail, une certaine exigence professionnelle, un sens de leur mission, une vision du service public.

obligatoirement comporter les motifs d'un éventuel préavis de grève. Le préavis doit, lui, être déposé cinq jours francs avant la cessation du travail. Enfin, un plan de prévisibilité d'entreprise définit les catégories d'agents indispensables

de transport défini par l'autorité organisatrice, qui est en première ligne avec les usagers. Allonger ce délai est utile pour limiter les perturbations dues aux grèves, sans porter atteinte de manière excessive au droit de grève.

à des services urbains ou suburbains et les lignes de fret locales utilisées par une seule entreprise ferroviaire, du champ d'application des règles relatives à la gestion des installations de service. Il reprend en réalité les dispositions de l'article 19 du projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français, article contre lequel notre groupe avait déjà voté. Si nous comprenons la volonté d'alléger les contraintes reposant sur les opérateurs ferroviaires de proximité, qui sont des entreprises ferroviaires locales, souvent des PME, assurant des services de fret de proximité et permettant ainsi l'acheminement des marchandises sur les premiers ou les derniers kilomètres,

rectificative en date du 20 février dernier, qui a privé les parlementaires des moyens effectifs de procéder à des auditions et d'examiner sérieusement ces mesures. Il y va ici des pouvoirs de contrôle du Parlement.

qui serait chargé à la fois de l'infrastructure et du service. Cela correspond à une vision extrêmement limitative et restrictive de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

du Gouvernement ? Contrairement à ce qui est mentionné dans l'exposé des motifs, il ne s'agit pas de dispositions qui auraient été subrepticement introduites à la dernière minute, puisque vous avez eu l'occasion de débattre de ces sujets lors de l'examen

-du champ d'application des règles de gestion des installations de service, conformément à une dérogation instruite par la directive 2012/34/UE. L'adoption de cette disposition permettra d'alléger les contraintes reposant sur les opérateurs ferroviaires de proximité, qui sont qui sont des entreprises ferroviaires locales, souvent des PME, assurant des services de fret de proximité et permettant ainsi l'acheminement des marchandises sur les premiers ou les derniers kilomètres. Elle permettra également à ces opérateurs de continuer d'assurer la gestion de lignes ferroviaires capillaires par délégation de SNCF Réseau et de participer ainsi au maintien d'une desserte fine des territoires.

évoluer. Les amendements prévoient la mise en place d'une palette de solutions pour une implication graduelle des régions en fonction de la réalité physique des lignes et du choix politique de chaque territoire. Le ministère des transports aura à se prononcer sur les options qui emportent la désignation d'un maître d'ouvrage autre que SNCF Réseau. Cette palette de solutions se décline en trois amendements : la mise en place de différents modèles, en dehors du transfert de propriété ; une solution complémentaire, transfert de propriété de lignes locales ou régionales à faible trafic à des collectivités locales ; l'exclusion du champ de la régulation par l'Arafer des lignes « verticalement intégrées », c'est-à-dire organisées sur le modèle du transport guidé- métro, tramway -sans séparation entre le gestionnaire d'infrastructure et l'exploitant de service. Le présent amendement est relatif à cette exclusion de certaines catégories de lignes, notamment les lignes strictement locales, du champ des dispositions habituellement applicables en matière de régulation.

permettre le transfert de la gestion des lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de son assemblée délibérante.

: La parole est à Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à rétablir la mission « accessibilité » de la SNCF au sein de l'EPIC de tête. Parmi les missions transversales devant être rattachées à SNCF Réseau figure la coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire. cette mission est dévolue à l'EPIC de tête SNCF. Il semble nécessaire de maintenir demain cette coordination au niveau de la holding de tête, c'est-à-dire au niveau de la future société nationale SNCF, plutôt que de la transférer à SNCF Réseau. le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau est responsable de la mise en accessibilité des quais. Demain, quand la gestion des gares de voyageurs aura été confiée à une filiale de SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure sera également responsable de la mise en accessibilité des gares de voyageurs, au bénéfice de l'ensemble des entreprises ferroviaires. Toutefois, les enjeux financiers considérables de la mise en accessibilité des infrastructures rendent encore plus nécessaire de concevoir, en parallèle, des services susceptibles de pallier le manque d'accessibilité de certaines parties du réseau, notamment La perspective de l'ouverture à la concurrence ne doit pas conduire à dégrader l'offre de mobilité proposée à ces publics sensibles. Il est donc nécessaire de maintenir au niveau de la société nationale SNCF la coordination des acteurs du groupe pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national bénéfice des personnes handicapées ou à mobilité réduite, cela sans préjudice des programmes de travaux d'accessibilité que SNCF Réseau mènera pour le compte de toutes les entreprises ferroviaires dans les gares de voyageurs et sur les quais et des dispositions que les autres opérateurs de transport

C'est notamment le cas des missions transversales, comme la gestion de crise et la coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transports ferroviaires au bénéfice des personnes handicapées ou à mobilité réduite. De telles missions devant être effectuées au bénéfice de l'ensemble des acteurs du transport ferroviaire-

Cet article vise à simplifier certaines règles et normes au bénéfice d'entreprises ferroviaires qui opèrent sur des lignes spécifiques, comme les lignes touristiques ou les lignes dédiées à des opérations de fret ferroviaire de proximité. Il exonère ces entreprises de l'obligation d'être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire.

par l'accès à une installation en fonction de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire. De plus, le règlement d'exécution de 2017 indique que ces installations font l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt pour être mises en crédit-bail ou en location. le Gouvernement prévoit donc de supprimer les autres cas dans lesquels le propriétaire peut ne pas donner suite à la manifestation d'intérêt du nouvel arrivant.

fait l'objet d'études ou de travaux en vue de maintenir la destination de l'infrastructure ; si le propriétaire, n'exploitant pas lui-même l'installation, décide d'en assurer lui-même directement l'exploitation.

Ces amendements tendent à réaffirmer la volonté du législateur d'assurer une mise en oeuvre à la fois rigoureuse et adaptée du principe de soutenabilité, lorsqu'il s'agit de services conventionnés.

Aujourd'hui, l'article L. 2221-8 du code des transports fixe l'obligation de détenir une licence pour assurer la conduite d'un train sur l'ensemble sur l'ensemble du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui y sont reliées, y compris les lignes d'accès aux installations de service et les lignes pouvant desservir plus d'un client final. Néanmoins, le dernier alinéa de l'article L. 2221-8 dispense de cette obligation les personnes « réalisant, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructure, des circulations limitées et à vitesse réduite sur le réseau ferroviaire au départ et à destination d'une voie non ouverte à la circulation publique qui lui est reliée

Pour obtenir cette licence, il faut satisfaire à certaines conditions de formation et de connaissances professionnelles. Il faut également justifier d'aptitudes physiques et psychologiques. La plupart du temps, ladite licence est également associée à des

des conducteurs qui n'ont pas vocation à circuler sur l'ensemble du réseau ferré européen : ils interviennent sur des infrastructures très locales, en particulier les réseaux séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire, destinés à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains, les infrastructures ferroviaires privées destinées à être exclusivement opérées par leurs propriétaires et des sections de voies temporairement fermées à la circulation.

Seule la fermeture administrative d'une ligne ou d'une section de ligne est encadrée par une procédure formalisée après consultation des parties, aux termes de l'article 22 du décret n° 97-444 Néanmoins, ces fermetures administratives n'interviennent que plusieurs années après la fin effective de la circulation des trains. Cet amendement vise donc à renforcer le le contrôle des acteurs intéressés, en particulier des régions, en transformant l'information en véritable consultation. Cela permettrait une véritable gouvernance partagée, afin de renforcer la transparence des décisions de fermeture à la circulation. Alors que la pérennité de nombreuses lignes du quotidien est remise en cause, l'adoption de cet amendement nous apparaît particulièrement nécessaire. Quel est l'avis de la commission ? Le droit en vigueur prévoit déjà que l'État et SNCF Réseau informent les régions de tous projets de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national, de tous projets de réalisation d'une nouvelle infrastructure ou d'adaptation de l'infrastructure existante, ainsi que de tous changements dans les conditions d'exploitation de ce réseau dans leur ressort territorial. Ces changements étant généralement motivés par des considérations de sécurité, il ne semble pas judicieux d'accroître le formalisme de ces procédures en les conditionnant à une décision du conseil d'administration ou de surveillance de SNCF Réseau. La commission

essayé d'améliorer, autant que faire se peut, ce texte dont chacun s'accorde à reconnaître l'importance, à la fois pour nos concitoyens, pour la mobilité et pour le développement durable.

très à l'écoute de nos demandes et qui s'est toujours montrée attentive à nos expressions, même lorsqu'elles étaient directes et franches. J'adresse aussi mes remerciements à l'ensemble de mes collègues de tous les groupes politiques : aussi bien en

inscrit un versement mobilité à taux réduit pour les EPCI qui n'ont pas de services réguliers de mobilité. Nous avons également mis en place un dispositif complémentaire de TICPE et fléché certains certificats d'économie d'énergie vers des actions en faveur de la mobilité propre.

Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs, afin de favoriser les mobilités dans les zones peu denses. Je pense notamment à l'optimisation des services de transport scolaire. M. Dantec

Le Sénat a voulu encourager le développement des véhicules à faibles émissions. Nous avons amélioré le dispositif du forfait mobilité durable en l'ouvrant aux conducteurs qui effectuent un trajet en covoiturage et en permettant le cumul de ce forfait avec le remboursement des frais de transport en commun, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Nous avons également permis aux employeurs de prendre en charge une partie des frais engagés par les salariés pour l'alimentation des véhicules électriques ou à hydrogène et adopté des dispositifs en faveur du verdissement des flottes

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous venons de vivre six jours de débat très riche sur le projet de loi d'orientation des mobilités.

Je salue également M. le président de la commission, l'ensemble des sénateurs qui se sont mobilisés sur ce texte, les administrateurs de la commission, dont je sais le professionnalisme et la rigueur, ainsi que l'ensemble des collaborateurs des groupes et des sénateurs qui ont travaillé sur ce texte.

et des priorités cohérentes : l'importance de l'entretien des infrastructures et des transports du quotidien est reconnue. Je souhaite remercier votre rapporteur, ainsi que l'ensemble des sénateurs, d'avoir respecté l'économie générale de ce volet,

salue en particulier l'adoption d'un plan d'action pour la mobilité solidaire et de mesures en faveur des personnes handicapées. Concernant les données et les nouvelles mobilités, je tiens